j’ai un sentiment étrange en présentant, pour la dixième année consécutive, le budget de la mission « Justice » : devons nous vraiment débattre comme nous le faisons chaque année, comme si la discussion du projet de loi de finances ne risquait pas de s’arrêter dès demain ? Oui, nous le devons, parce que c’est l’une des missions les plus essentielles des parlementaires que de discuter et de voter le budget. Nous le devons aussi parce que, même si tout s’interrompait demain, il faudra bien que le débat reprenne ultérieurement afin de doter la France d’un budget pour 2025. Le Sénat pourra alors s’appuyer sur le travail déjà réalisé et consacré par les votes exprimés en séance publique depuis huit jours sur la première partie de la loi de finances et sur les premières missions budgétaires de la seconde partie. Il me paraît donc crucial que, malgré le nombre élevé d’amendements, nous ne dépassions pas les délais ce soir et que nous allions jusqu’à l’adoption des crédits de la mission « Justice ». En effet, nous ne pouvons pas dire non à un budget qui est en hausse de 108 millions d’euros, hors contribution aux pensions et à périmètre constant, et pour lequel le Gouvernement propose une augmentation supplémentaire de 250 millions d’euros, au moment même où la situation budgétaire contraint la plupart des ministères à des économies. Les politiques de la justice elles mêmes ont été fortement affectées par les économies en 2024, le décret d’annulation du 21 février, suivi de surgels de crédits, ayant causé de réelles difficultés de gestion – je pense notamment aux renouvellements de contrats dans la protection judiciaire de la jeunesse En 2025 également, ce budget reste en retrait par rapport à ce que prévoyait la loi de programmation ; des choix devront être faits. La priorité est donnée à la poursuite de l’augmentation des moyens humains, avec la création de 619 postes, dont 270 pour les services judiciaires. La progression des moyens est donc préservée, mais reste inférieure au rythme prévu par la loi de programmation. Dans l’administration pénitentiaire, les nouveaux surveillants seront affectés exclusivement aux nouveaux établissements : il ne s’agit pas d’un surplus dans les établissements existants. Cette augmentation des effectifs s’appuie sur une politique de revalorisation des métiers, indispensable pour attirer et retenir les personnels, notamment les magistrats, les greffiers et les personnels de l’administration pénitentiaire.

la création de 15 000 places n’est pas un luxe : elle permettra tout au plus de contenir l’inflation du nombre de détenus et la surpopulation carcérale. La poursuite du plan « 15 000 places de prison », même avec une échéance décalée à 2029, reste et doit rester une priorité. Toutefois, je plaide pour une plus grande standardisation des programmes, ainsi que pour un pilotage plus efficace, qui associe les personnels en amont, car j’ai constaté trop de malfaçons dans les établissements livrés. La plupart de ces observations valent aussi pour le programme de construction de vingt centres éducatifs fermés. Les autres dépenses sont soumises à de fortes restrictions. Je m’inquiète notamment pour la modernisation de la fonction informatique. L’obsolescence de nombreux applicatifs est une difficulté importante, au quotidien, pour les magistrats et pour leurs équipes obère leur capacité à répondre aux attentes – légitimes – des citoyens, qui appellent de leurs vœux un service public de la justice efficace et rapide. La sécurisation des locaux, en particulier dans les prisons, à la suite de l’attaque d’un fourgon en mai dernier, ne saurait, en revanche, être mise de côté pour des raisons budgétaires. Des quantités invraisemblables de téléphones et autres produits sont livrés par drones, et les services des prisons peinent à lutter contre ce phénomène. L’effort doit être poursuivi et, de manière générale, les engagements pris auprès des personnels en matière de sécurisation devront être tenus. Toutefois, je suis particulièrement préoccupé par la progression considérable des frais de justice, qui seront passés de moins de 500 millions d’euros en 2017 à près de 750 millions d’euros en 2025. Que ce soit sur les frais de gardiennage ou sur les demandes d’expertise, une réflexion d’ampleur est nécessaire, en lien avec les services d’enquête de la police et de la gendarmerie. Je comprends bien la nécessité de participer à l’effort collectif de redressement des finances publiques. Il convient cependant de rappeler quelle crise profonde traverse le monde de la justice et le service public de la justice dans notre pays, crise rappelée lors des États généraux de 2021 et constatée par tous nos concitoyens qui ont recours des politiques de l’État les plus anciennes et les plus fondamentales. Elle a souffert de décennies d’oubli, que l’accroissement actuel des moyens ne compense que très partiellement. La justice française dispose ainsi du plus faible budget par habitant en pourcentage du PIB parmi les pays de richesse comparable en Europe, et les délais sont dans notre En conclusion, mes chers collègues, la commission des finances vous propose d’adopter les crédits tels que prévus dans le texte initial du projet de loi et modifiés par les amendements du Gouvernement. Ces amendements permettront en effet, sans exonérer le ministère de la justice des efforts budgétaires nécessaires, de réaliser une part importante de la trajectoire prévue par la loi de programmation

l’administration pénitentiaire connaît une crise sans précédent, liée à la surpopulation carcérale, à l’inadéquation du nombre de postes et à l’emprise de plus en plus marquée de la criminalité organisée.

Nous saluons ces engagements et cette lucidité, raison pour laquelle la commission des lois a approuvé le budget du programme « Administration pénitentiaire ». Toutefois, le budget 2025 aurait dû être l’occasion de choix plus stratégiques. doit être de réorienter les crédits des projets immobiliers pour améliorer plus rapidement les conditions de détention et les conditions de travail des personnels.

plus de deux fois supérieur à celui des personnes détenues. C’est donc là qu’il faut agir ! Or les crédits alloués aux missions en milieu ouvert sont en légère décroissance, confirmant une moindre attention portée à ces actions, dont l’administration pénitentiaire et les acteurs de terrain soulignent pourtant tous le caractère indispensable. Les mesures de milieu ouvert sont trop souvent vues comme des alternatives à l’incarcération, ce qui est tout à fait faux : ce sont des mesures spécifiques, qu’il faut prendre pour elles mêmes.

Une revalorisation du milieu ouvert, notamment l’évaluation et le développement des mesures de suivi, est indispensable à court terme, pour lutter contre la surpopulation carcérale, et, plus fondamentalement, pour permettre le prononcé de peines socialement utiles.

voilà plusieurs années que la situation du ministère de la justice suscite notre plus vive préoccupation, laquelle explique l’attachement du Sénat à la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice pour les années 2023 à 2027, la fameuse LOPJ. Ce texte porte l’ambition de remédier au manque chronique de recrutement et d’investissement de la Chancellerie et ainsi de restaurer la qualité des conditions de travail des agents judiciaires, donc, par là même, le bon fonctionnement de la justice.

conduirait à renoncer aux objectifs de recrutement et à abandonner de nombreux investissements, notamment immobiliers et numériques. Les crédits consacrés à l’immobilier judiciaire et à l’informatique ministérielle diminueraient ainsi respectivement et de 37 millions d’euros par rapport à la loi de finances 2024. La commission des lois a donc accueilli avec une grande satisfaction, monsieur le garde des sceaux, votre annonce du 31 octobre dernier. L’arbitrage budgétaire que vous avez obtenu permettrait, d’une part, de respecter la trajectoire de recrutement établie en LOPJ, grâce à la création de 343 postes de magistrats, de greffiers et de 307 postes d’attachés de justice, et, d’autre part, de préserver les investissements immobiliers et numériques du ministère, auxquels seraient respectivement alloués 47,4 millions et 49 millions d’euros. La commission se réjouit que, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, l’essentiel soit sauf. Nous sommes en effet attachés à ce que la situation de la justice s’améliore, même dans pareil contexte. Il serait utile, à cette fin, que les services de la Chancellerie continuent de travailler à réduire le dynamisme de certaines dépenses qui grèvent significativement son budget. La commission s’intéresse particulièrement au plan de maîtrise des frais de justice. Ces frais ont connu une hausse drastique ces dernières années ; il est impératif de les contenir. Le plan de maîtrise commence à porter ses fruits. Ainsi, la croissance du coût des mémoires déposés fléchit peu à peu elle était de 12 % entre 2020 et 2021 ; elle se limite à 5 % entre 2023 et 2024. Il faut poursuivre cette dynamique. Les objectifs que vous avez identifiés pour 2025, à savoir la réduction de 20 % des coûts du gardiennage de véhicules et le développement du recours à la (Pnij), devraient le permettre. Une autre piste a été avancée : celle de la modulation de l’aide juridictionnelle, grâce à deux mesures spécifiques,

intervention et confirme qu’à nos yeux il est primordial de préserver trois politiques du ministère pour rétablir les conditions de travail des agents et restaurer le bon fonctionnement de la justice : il s’agit, sans surprise, du recrutement, du numérique et de l’immobilier.

Par rapport au nombre d’inscrits, le nombre de greffiers réellement recrutés est faible ! La commission a été attentive, à cet égard, à l’application des accords du 26 octobre 2023. Nous suivrons avec intérêt les travaux de la Chancellerie quant à l’organisation des juridictions, qui mérite d’être précisée afin que chacun y trouve sa place. L’attractivité des professions judiciaires repose évidemment, par ailleurs, sur les politiques numérique et immobilière du ministère. la commission demeure préoccupée par la maintenance et le développement des applicatifs numériques de la Chancellerie, car le mécontentement des personnels perdure. Nous suivrons donc avec attention le travail du ministère à ce sujet, qu’il s’agisse de la réduction des trames du logiciel Cassiopée ou de l’expérimentation puis de la mise en œuvre progressive de Portalis, dont nous parlons depuis déjà quatre ans. La politique immobilière, enfin, suscite l’inquiétude de la commission. La situation budgétaire que nous traversons affecte particulièrement l’immobilier judiciaire, car de tels projets nécessitent de la prévisibilité financière. Nous en manquons actuellement, et il est urgent d’y remédier. Je ne suis, hélas ! pas certaine que nous y Au delà, si la politique de consultation du ministère semble bien structurée, il importe de veiller à ce qu’elle ne soit pas strictement formelle, les personnels s’estimant peu entendus sur ces sujets.

fait notamment d’une augmentation de la charge de travail depuis la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs, qui est une bonne chose, mais dont l’effet

182. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir.

et de programmation du ministère de la justice, votée pas plus tard que l’an dernier, prévoit un renforcement, qui est à la fois nécessaire et urgent, du budget de ce ministère régalien, qui a trop longtemps souffert d’un sous investissement chronique. Elle prévoit notamment la création de 1 500 postes de magistrats, de 1 800 postes de greffiers et de 1 100 postes d’attachés de justice d’ici à 2027. Il y a donc de quoi être déconcerté en découvrant que près d’un demi milliard d’euros manquent à l’appel dans le budget initial de la mission « Justice » du projet de loi de finances, d’autant que cette baisse des crédits par rapport aux objectifs fixés doit aussi s’apprécier à l’aune des annulations décidées par décret en février dernier. la contrainte budgétaire est ce qu’elle est. Mais, comme le ministre de l’intérieur nous le rappelait encore hier soir, un budget, ce ne sont pas que des chiffres ! Ce sont surtout des choix politiques. Aussi me semble t il primordial de saluer l’effort du garde des sceaux, qui a réussi à obtenir un arbitrage favorable. Celui ci nous permettra de voter, tout à l’heure, un abondement de près de 250 millions d’euros en faveur de la mission, qui bénéficiera,, de 924 ETP supplémentaires.

La baisse majeure prévue pour les crédits du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » sera quant à elle finalement limitée. Pour autant, cette évolution ne représente aucunement un investissement dans notre institution judiciaire, qui en a pourtant grandement besoin. Je veux rappeler les chiffres établis par la Commission européenne dans son dernier rapport – nous les connaissons bien, mais il est essentiel d’y insister. La France compte 11,3 juges pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de 21,9.

Comment peut on imaginer que la justice puisse être rendue dans des délais raisonnables et dans de bonnes conditions avec si peu de magistrats professionnels ? Nous dépensons à peine 0,2 % de notre PIB pour la justice, quand la majorité de nos voisins en dépense 0,3 La présentation du budget pour 2025 doit donc être analysée dans ce contexte de délabrement et de souffrance pour tous les professionnels, souffrance largement partagée par de nombreux magistrats et greffiers, mais également subie par les auxiliaires de justice. Cette souffrance n’est pas abstraite quatre greffiers se sont donné la mort cette année. Et je n’apprends à personne que cette absence de moyens touche tous les services ! Prenons l’exemple du juge des enfants. La France en compte 522. Il en faudrait 235 de plus, d’après le Syndicat de la magistrature, d’autant qu’un tiers de ces juges tiennent leurs audiences sans greffier. Cette charge de travail affecte forcément le suivi des situations et la qualité de la préparation des décisions rendues. Nous revenons donc de très loin, et ce budget ne permettra pas de combler le retard.

dans les années qui viennent. L’utilisation de l’intelligence artificielle augmente et augmentera les recours déposés, alors que notre justice ne semble pas encore tout à fait outillée pour répondre à ce nouveau défi ; une mission d’information de la commission des lois travaille actuellement sur ce sujet.

Enfin, même lorsque les crédits de paiement sont à la hausse, comme pour le programme « Administration pénitentiaire », l’effort n’est pas suffisant. Le garde des sceaux a lui même reconnu dernièrement que les objectifs du « plan 15 000 » ne seront pas tenus. Notre politique carcérale continue d’être obnubilée par les places de prison, alors que nous n’arriverons jamais à en construire suffisamment pour combler les besoins.

Nul ne peut ignorer non plus que, demain, à la même heure, notre gouvernement pourra avoir été renversé par une majorité plus qu’hétéroclite de députés. Notre Constitution n’a pas prévu que les sénateurs interviennent dans le processus conduisant à voter la censure du Gouvernement.

Ce travail au long cours, mis en regard d’une certaine instabilité gouvernementale, permet à notre chambre de conserver une vision indispensable à une meilleure justice pour demain, au service de toutes

d’euros, soit 2 % de crédits de paiement supplémentaires. S’il correspond à une stagnation des moyens en euros constants, ce montant permet une poursuite des chantiers engagés. Il faut encore saluer, monsieur le garde des sceaux, l’arbitrage, dont d’autres ont parlé avant moi, que vous avez obtenu. Cet arbitrage se traduit par un abondement de 250 millions d’euros supplémentaires, qui permettra de préserver le schéma de recrutement de votre ministère et l’essentiel de ses investissements numériques. À ce sujet, j’ai noté, comme vous, mes chers collègues, la possibilité ouverte aux victimes de certaines atteintes aux biens de porter plainte en ligne. En tant que sénatrice des Français de l’étranger, j’espère que cette faculté sera prochainement accessible à nos ressortissants français à l’étranger, particulièrement en cas d’atteinte aux personnes. Cette possibilité pourrait être extrêmement profitable aux victimes de violences intrafamiliales (VIF) à l’étranger, dont l’éloignement rime avec isolement. L’effort budgétaire, qui était indispensable, doit être poursuivi. Si les moyens de la justice ont crû de 36 % depuis 2020, nous devons aller encore plus loin pour atteindre les standards européens les pays comparables à la France consacrent à la justice, en moyenne, 92,10 euros par habitant, contre 77,20 euros pour notre pays. Les enjeux sont considérables s’agissant d’un pouvoir régalien, qui est un ciment pour notre société. Si la justice, par essence, exige temps et impartialité, elle ne doit pas être perçue comme lointaine et indifférente ; nous ne saurions laisser s’installer un fossé entre l’institution et celles et ceux qu’elle sert. C’est pourquoi il est indispensable que la justice judiciaire accompagne les évolutions de la société, dont les grands procès sont un marqueur.

permet à chacun de s’interroger sur les monstres ordinaires qui peuplent notre société. Une autre affaire médiatisée, dite de Julie, lui fait écho : cette mineure de 13 ans, affaiblie par une maladie chronique, a été abusée par des pompiers dans des proportions qu’il appartient à notre système judiciaire de Ces deux dossiers illustrent, si besoin était, la difficulté d’appréhender la notion de consentement. Alors que la commission des lois et la délégation aux droits des femmes travaillent ensemble, ce qui est à saluer, sur la prévention de la récidive, je note les initiatives parlementaires, dans nos deux chambres,

de profondément absurde à discuter de ce budget alors même que tout le monde sait le sort qui vous sera réservé demain, monsieur le garde des sceaux. On n’en sait que ce gouvernement vit ses dernières heures. Absurde, parce que tout le monde sait que ce gouvernement perdra, demain, la dernière once de légitimité qui lui restait. Alors taisez vous ! Absurde, parce que ce scénario était au fond écrit d’avance. Il est absurde aussi d’imaginer que l’on puisse diriger un pays comme la France en tournant à ce point le dos au verdict des urnes ; absurde encore de continuer, les uns et les autres, les unes et les autres,

que nous débattons d’un texte budgétaire présenté par ce gouvernement en fin de vie. Et nous ne pouvons de nouveau que souligner nos désaccords profonds avec votre politique. Le budget que vous nous présentez continue de sous

en Allemagne, soit plus du double ! Or, derrière ces chiffres et sous les crédits que nous votons aujourd’hui, c’est bien notre État de droit qui est en jeu, porté à bout de bras par nos professionnels de la justice. Ceux ci nous le rappellent fréquemment, au travers des mouvements sociaux. L’exemple récent, déjà mentionné, du mouvement de grève des agents de la PJJ est à cet égard éloquent. C’est à la suite de l’annonce du non renouvellement de 500 agents contractuels que ces professionnels nous ont alarmés sur la situation catastrophique du secteur. Ils nous ont rappelé l’épuisement de ces travailleurs, déjà en sous effectif. La droite et l’extrême droite ne cessent de vouloir punir toujours davantage les mineurs délinquants. Pourtant, l’accompagnement des jeunes en difficulté est particulièrement altéré par la saturation des établissements et des services. Les éducateurs, les psychologues, les assistants sociaux et les personnels administratifs sont surchargés, mais ni solutions ni moyens ne leur sont octroyés. Je voudrais aussi souligner que ce budget ne respecte pas les objectifs de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027. Il avait pourtant été annoncé qu’elle permettrait de rattraper plus de trente ans d’abandon budgétaire, politique et humain de notre justice. À peine votée, cette loi est d’ores et déjà obsolète ! Au fond, tout cela montre à quel point nous avons besoin, dans ce domaine comme dans d’autres, d’un changement de politique ; il est à souhaiter qu’il arrive le plus vite possible.

de Fresnes… « La justice est la vérité en action. » Victor Hugo nous rappelle que l’exercice judiciaire n’est pas seulement une affaire de lois, mais aussi une quête de sens, un engagement envers la dignité humaine et l’équité sociale. Or, en France, notre système judiciaire peine à incarner ces principes. Malgré les efforts budgétaires engagés, la surpopulation carcérale reste un fléau, avec 80 000 personnes en détention. Le taux d’occupation dépasse 140 % dans certaines maisons d’arrêt, et des milliers de détenus sont contraints de dormir sur des matelas à même le sol. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques : ils traduisent une réalité indigne et des échecs structurels. Le choix de construire toujours plus de prisons est à cet égard une fuite en avant ces investissements massifs ne résolvent pas le problème. Entre 1990 et aujourd’hui, nous avons augmenté nos capacités carcérales de plus de 24 000 places, sans pour autant enrayer la surpopulation ou améliorer les conditions de détention. Pis, chaque nouvelle place semble rapidement occupée, confirmant que nous privilégions une logique punitive au détriment de la prévention. Nous devons changer de paradigme. Une société juste ne peut reposer sur une surenchère pénale qui stigmatise les plus vulnérables. En effet, qui retrouve t on en prison ? Des hommes et des femmes jeunes, souvent sans diplôme, précaires, dont plus de 40 % ont subi des violences dans leur enfance. La prison crée un cercle vicieux de désocialisation et de récidive

La justice que nous défendons ne se limite pas à punir : elle respecte la dignité de chacun et vise à réparer, à réinsérer et à prévenir. Monsieur le garde des sceaux, trois axes doivent guider notre action. Premier axe : comprendre et humaniser la peine. Celle ci ne doit pas être une abstraction : elle doit être expliquée, comprise et adaptée à la personne condamnée, aux victimes et à la société. Cela passe par une meilleure éducation, dès le plus jeune âge, sur le fonctionnement de la justice, mais aussi par l’accompagnement des victimes et par la promotion de la justice restaurative. Deuxième axe : investir dans des alternatives crédibles à la détention. Le recours à la prison doit être l’exception, et non la norme ! Nous devons généraliser les peines de probation, les placements extérieurs et les travaux d’intérêt général, tout en assurant un accompagnement socio éducatif solide. Cela nécessite des moyens humains, des magistrats, des éducateurs, des médiateurs. Les comparutions immédiates, qui favorisent des décisions hâtives et trop souvent répressives, doivent être limitées.

Nous devons réduire drastiquement la détention provisoire, respecter les normes internationales d’encellulement individuel et assurer un accès effectif aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation ou de l’emploi. Chaque détenu sortira un jour. Notre responsabilité est de préparer cette sortie pour éviter que la prison ne soit qu’un temps perdu, destructeur pour l’individu et dangereux pour la société.

Sans ressources, monsieur le garde des sceaux, toutes les réformes resteront lettre morte. Mes chers collègues, la justice ne peut être réduite à une simple comptabilité des crimes et des peines : elle est une institution essentielle de notre démocratie, qui doit protéger les libertés, réparer les torts et préparer l’avenir.

mais aussi d’une juridiction spécialisée dans le traitement des violences intrafamiliales, combat que je mène depuis longtemps et qui a été en partie satisfait par les travaux de Dominique Vérien, lesquels ont permis l’émergence des pôles spécialisés.

c’était en octobre 2023 : le Sénat adoptait les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027. Les objectifs étaient ambitieux : réformer certains champs de notre justice pour la rendre « plus rapide, plus claire, plus moderne Les moyens l’étaient également : entre 2023 et 2027, le budget du ministère devait augmenter de 21 %. C’était en octobre 2023. Nous avions l’espoir que ce grand service public de la justice serait restauré après des années de disette, quel que soit le Gouvernement. un an plus tard, à l’aune des contraintes financières qui encadrent les débats sur le projet de loi de finances de notre pays, cette dynamique est interrompue. En effet, si les crédits sont maintenus par rapport à l’an dernier, à 10,2 milliards d’euros contre 10,1 milliards en 2024, ils sont en deçà des 10,7 milliards d’euros prévus par la loi de programmation. Nous saluons l’inflexion du Gouvernement, qui nous rapproche de l’exécution budgétaire prévue, mais nous ne pouvons pas accepter que la trajectoire ne soit pas respectée, car cela se fait au détriment de la justice.

Le groupe Les Indépendants a toujours défendu la réduction de la dépense publique, mais non de n’importe quelle dépense publique. En effet, seul l’État est en mesure d’exercer les missions régaliennes, qui sont au fondement du fonctionnement de notre société et au cœur des demandes de nos concitoyens. Ce budget n’est pas celui de la reconstruction et de la projection qu’attendent les acteurs du monde judiciaire. La justice, la police, les armées ou encore l’enseignement supérieur et la recherche ne sauraient en aucun cas pâtir des difficultés budgétaires que notre pays rencontre actuellement. Comment allons nous expliquer à nos concitoyens que la justice, sur laquelle ils comptent pour faire valoir leurs droits, va encore devoir attendre ? souligne que la justice française dispose du plus faible budget par habitant, en pourcentage de PIB, de l’ensemble des pays comparables. Tous les orateurs l’ont rappelé ici ce soir : le retard est structurel. Combien de temps accepterons nous encore d’avoir une justice sous dotée, alors que des marges financières importantes on le sait, au sein des autorités administratives indépendantes ou des opérateurs de l’État ? Ce n’est pas notre collègue Nathalie Goulet qui me contredira.

Il est possible de trouver auprès des autorités administratives indépendantes des marges bien supérieures aux 276 millions d’euros qui manqueront à la justice

Mais il faut donner à la justice les moyens de poursuivre une modernisation qui vient à peine de commencer. Or les solutions informatiques dont dispose le ministère sont pour le moins insuffisantes. La restauration de la justice doit demeurer l’un des chantiers prioritaires des prochaines années : il y a là une attente

L’efficacité de la justice passe aussi par des moyens modernes. Tout le monde a fait valoir, à juste titre, combien le plan numérique n’avait

en réalité, elle n’inspire plus aucune confiance aux citoyens. Lorsque nous parlons de la justice, au delà de ce grand service public régalien, c’est donc de notre système d’État de droit, dans lequel la démocratie peut

la mission « Justice » porte en elle l’essence du régalien, tout en ayant l’ambition d’accompagner les justiciables au plus près de leurs réalités quotidiennes. ligne de la trajectoire budgétaire engagée depuis 2017, cette mission connaît une nouvelle progression : son enveloppe de 12,46 milliards d’euros en crédits de paiement est en hausse de 108 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

Les priorités fléchées en 2025 auront notamment pour effet d’améliorer les délais de traitement des décisions de justice et de renforcer le soutien des juridictions judiciaires, en poursuivant les projets d’immobilier judiciaires, qui permettront d’accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux effectifs.

À ce titre, l’aide juridictionnelle constitue la majeure partie des crédits de ce programme, sans oublier l’accès au droit, qui reste fondamental. L’ambition demeure, à cet égard, de faire reculer les zones de non droit et de combattre la peur, l’illettrisme et l’illectronisme. C’est pourquoi je souhaite renforcer le financement des bus itinérants. Il est indispensable d’amener la justice au plus près des campagnes françaises, notamment en outre mer. Ce renforcement de l’accès aux droits permettra aux femmes victimes de violences de continuer à bénéficier, par exemple, des téléphones grave danger, dont plus de 6 000 étaient déployés en juillet 2024, ce qui est considérable.

rupture de parcours. Par ailleurs, 4 millions d’euros seront consacrés à la construction de nouveaux centres éducatifs fermés, pour augmenter notre capacité d’accueil de ce public particulier.

Les défis pour cette administration sont de taille, et les objectifs pour 2025 contribueront à y faire face. Je pense tout d’abord au renforcement de la sécurité des personnels et des structures pénitentiaires, indispensable après le drame d’Incarville, au

la formation professionnelle et les activités en détention. Enfin, il faut améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires qui sont confrontés à la surpopulation carcérale chronique.

Sur ce point, au regard de l’accroissement constant de la pression carcérale, il est évident que le seul programme immobilier ne suffira pas à endiguer durablement ce phénomène. Nous espérons tout de même que la poursuite du « plan 15 000 » permettra d’apporter une solution.

Pour concrétiser tous ces engagements, des recrutements massifs sont indispensables. Les crédits alloués à la justice pour 2025 permettront l’embauche de nouveaux magistrats, greffiers, attachés de justice, agents pénitentiaires et éducateurs de la PJJ. Alors que le projet initial prévoyait une baisse de 500 millions d’euros, nous nous réjouissons des ajustements budgétaires récemment annoncés, qui permettront de respecter les engagements de la LOPJ. Bien conscient des contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur cette mission, mais également des efforts qui ont été accomplis pour maintenir nos compatriotes au cœur de ce service public,

Je tiens donc à aborder la situation du PNF. Le parquet national financier, dont le budget relève du programme 166, n’est pas mentionné dans le document de politique transversale sur la fraude et l’évasion fiscales. C’est une carence.

souligné, je concentrerai mon propos sur le programme 182, « Protection judiciaire de la jeunesse ». Chacun sait l’importance de ce programme consacré aux mesures éducatives et judiciaires destinées aux mineurs et aux jeunes adultes, et sa place dans notre dispositif judiciaire.

des contraintes budgétaires et des problématiques liées aux ressources humaines. Contrairement aux autres acteurs de la justice, la PJJ n’a pas connu d’augmentation significative de ses moyens à la suite de la loi d’orientation et de

mesdames, messieurs les sénateurs, je suis devant vous ce soir pour débattre du budget pour 2025 du ministère de la justice. Comme vous le savez, le projet de loi de finances constitue, pour l’ensemble des gens de justice – magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, fonctionnaires et agents des services judiciaires de l’administration pénitentiaire et de la protection de la jeunesse –, mais aussi, et surtout, pour l’ensemble de nos concitoyens, le marqueur de la force et de la réalité de nos engagements en matière de justice dans notre pays. Cela ne va pas durer ! À ce titre, le projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier en conseil des ministres, fondé sur la lettre plafond adressée à mon prédécesseur, a notamment été rehaussé

C’est la référence de tous les acteurs du monde judiciaire et, au delà des seuls professionnels de la justice, celle des élus nationaux et locaux, ainsi que de nos concitoyens.

mais aussi immobiliers. Ces demandes, auxquelles nos concitoyens sont fortement sensibles, sont indispensables à la réduction des délais de jugement et à la confiance dans la justice. C’est pourquoi, ainsi que le Premier ministre s’y était engagé, le ministère de la justice fait l’objet d’un effort significatif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, à hauteur de 250 millions d’euros supplémentaires par rapport à la lettre plafond. Le budget de la justice qui vous est présenté est donc rehaussé à 10,5 milliards d’euros, à la hauteur des engagements pris. L’allocation de 250 millions d’euros

Cet effort n’aurait pas été possible sans l’arbitrage favorable du Premier ministre et le soutien du ministre chargé du budget et des comptes publics, auxquels je renouvelle mes remerciements. un signal fort en faveur de la réparation de notre justice, alors que cette mission régalienne fondamentale a été trop longtemps délaissée. Entre 2024 et 2025, les crédits du ministère augmentent ainsi de 358 millions d’euros. Ces moyens sont importants. Vous le savez, je suis prioritairement attaché à maintenir les engagements pris sur les effectifs, condition pour parvenir à désengorger les tribunaux dont les délais d’audiencement sont devenus Il faut donc poursuivre les recrutements entamés à la suite des États généraux de la justice, à partir des moyens obtenus par mon prédécesseur, en les conjuguant à des mesures catégorielles ciblées, afin de renforcer l’attractivité des métiers de la justice. Ainsi, concernant l’année 2025, une autorisation de recrutement de 1 543

Par ailleurs, l’attention aux personnels et aux conditions de travail est un engagement fort de la loi d’orientation et de programmation, tout comme la garantie de l’attractivité des rémunérations des métiers de la justice. Grâce au rehaussement du budget, nous sommes

L’efficacité dans l’exécution des peines et l’accélération des procédures pénales font également partie des priorités. À ce titre, rien ne pourra se faire si nous n’avons pas la capacité de prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en particulier les personnes détenues, dans le respect et la dignité dus à chacun. C’est pourquoi j’insiste sur l’importance des crédits dédiés à la réhabilitation et à la maintenance au moins autant que sur celle des moyens alloués à la construction. Concernant la programmation immobilière pénitentiaire, les crédits dévolus en PLF pour 2025 sont conçus pour permettre la poursuite du plan de construction de 15 000 places supplémentaires. Je tiens à rappeler ici les difficultés que nous rencontrons dans le calendrier de réalisation des grandes opérations de construction. Ainsi, la réalisation du « plan 15 000 » est en retard moins d’un tiers est réalisé aujourd’hui, et 42 % seulement le seront d’ici à 2027. Ces difficultés sont liées à des facteurs exogènes indépendants de la volonté du ministère, qui ne sont toujours pas d’ordre budgétaire, comme des aléas techniques et environnementaux, des tensions générées sur les délais d’approvisionnement par les différentes crises ou la fragilité du tissu économique. Je le dis aussi sans détour devant la Haute Assemblée, qui est celle des territoires de la République : il est très souvent difficile de convaincre les élus de nous laisser bâtir un établissement pénitentiaire sur leur territoire. même été élu local. Je peux parfaitement le comprendre et je ne réduis pas nos difficultés à ces seules réticences. L’achèvement du « plan 15 000 » ne sera pas possible opérationnellement avant 2029 dans le meilleur des cas, et, au delà des accords que nous devrons obtenir des élus, cela supposera des efforts budgétaires substantiels dans les prochaines années. Il nous faut agir sur l’ensemble des leviers. C’est ce que j’ai demandé à Laurent Ridel, inspecteur général de la justice et ancien directeur de l’administration pénitentiaire, en lui confiant une mission d’accélération du programme pénitentiaire. Il nous faut en effet aller plus vite, en proposant

Ces mesures auront, nous l’espérons, un premier effet d’ici à 2027 sur l’augmentation du nombre de places livrables à cette échéance. Elles serviront aussi, et surtout, après cette date, car la construction ne s’arrêtera pas là. pas là. Mais encore une fois, rien ne sera possible sans la solidarité des élus autour de cette ambition, qui est aussi une cause de solidarité nationale. Concernant l’immobilier judiciaire, le budget proposé doit nous permettre de couvrir les opérations d’ores et déjà en chantier et de poursuivre la mise à niveau du parc immobilier, notamment au regard de la sécurité des personnes, des mises aux normes réglementaires, de la mise en sûreté des palais de justice et des opérations de gros entretien indispensables à la pérennité du patrimoine.

je souhaite mettre en lumière certaines enveloppes qui ont pour vocation de moderniser et d’améliorer concrètement le fonctionnement du service public de la justice, ainsi que les conditions de travail

progressivement de rattraper notre retard. En outre, les crédits consacrés aux techniques d’enquêtes numériques judiciaires sont portés à 49 millions d’euros. Ces crédits ont été calibrés pour permettre de poursuivre la dématérialisation et la modernisation de bout en bout de nos chaînes judiciaires civiles et pénales, avec la procédure pénale numérique, le projet de refonte civile Portalis, la dématérialisation complète du casier judiciaire national, la mise en convergence de nos outils applicatifs pénaux, ou encore le nouveau système d’information de l’application des peines Prisme. Les crédits de l’accès au droit et à la justice sont portés à 802 millions d’euros pour 2025, contre 790 millions d’euros en 2024. Plus spécifiquement, dans cette enveloppe, les crédits dédiés à l’aide juridictionnelle augmentent en 2025, pour atteindre 718 millions d’euros, soit 6 millions d’euros supplémentaires sur une année. Parallèlement, l’aide aux victimes est portée à 51 millions d’euros en 2025, soit une hausse de 4,5 millions d’euros par rapport à 2024. Sur ce point, je souligne que l’aide aux victimes de violences intrafamiliales constitue désormais 37 % du budget dévolu aux victimes. L’effort et l’organisation mis en place ces dernières années se poursuivront. Enfin, concernant l’action sociale offerte par le ministère à ses agents, action qui est essentielle pour assurer leur soutien et contribuer à l’attractivité de notre institution, le projet de budget prévoit la mobilisation de plus de 36 millions d’euros, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024. Plusieurs d’entre vous ont évoqué la fin de gestion 2024. Je suis parfaitement conscient des contraintes budgétaires considérables auxquelles nous sommes confrontés. Je suis attaché comme vous à la crédibilité financière de notre pays. Tout au long de l’exercice budgétaire 2024, mon ministère a pris part à l’effort budgétaire rendu nécessaire par la situation des finances publiques. Dans ce contexte, les efforts sur le fonctionnement consentis par mon ministère n’ont pas manqué de provoquer des mouvements sociaux

Le Gouvernement a ainsi accepté de réduire d’environ la moitié le montant des régulations successives de l’année. Ce geste prend en compte, d’une part, les efforts de maîtrise réalisés et, d’autre part, la nécessité de récupérer la nécessité de récupérer le quantum de crédits nécessaires au fonctionnement du service public de la justice d’ici à la fin de l’année, sans entraîner d’importants reports de charges obérant la gestion 2025.

L’enveloppe de crédits consacrée à cette action est portée à 748 millions d’euros. Cette dotation est en hausse de 11 % par rapport à 2024. À ce titre, et en sus du plan de maîtrise lancé en 2023, qui commence à porter ses fruits,

Au delà, conformément à l’organisation de nos travaux décidés par la conférence des présidents et en accord avec la commission des finances, la suite de l’examen de cette mission serait reportée au samedi 7 décembre

Grâce à la dernière loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la procédure pénale a été simplifiée et améliorée. En parallèle, jamais autant de moyens n’avaient été investis dans ce grand service public. Pour assurer la politique ambitieuse défendue par les gouvernements qui se sont succédé depuis 2017, il est indispensable de revaloriser les personnels en place, de recruter et de former massivement de nouveaux effectifs de magistrats, greffiers, assistants de justice et personnels pénitentiaires. notre amendement permettra de maintenir les engagements essentiels, notamment sur les recrutements. La

l’avis du Gouvernement ? La politique volontariste menée en la matière depuis plusieurs années et renforcée avec le Grenelle des violences conjugales a, je le crois, amélioré la situation. Parmi les mesures récentes, citons l’augmentation du recours aux réponses rapides, le développement de l’éviction du conjoint, l’ordonnance de protection, le téléphone grave danger mis à disposition des victimes, ou encore le bracelet antirapprochement. Par ailleurs, comme vous le savez,

permettent une action coordonnée et rapide de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, mais aussi des partenaires extérieurs concernés par une même situation familiale. Ils facilitent le partage d’informations et une plus grande articulation entre les procédures civiles et les procédures pénales engagées à l’encontre des conjoints ou parents violents. Si les efforts doivent évidemment être poursuivis, il convient de relever que la politique de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales ne relève pas de la seule institution judiciaire. Par ailleurs, il est à craindre que la création de juridictions spécialisées n’éloigne de nombreuses victimes du lieu de la réponse judiciaire, puisqu’il n’apparaît pas envisageable de créer des juridictions spécialisées au niveau de chaque tribunal judiciaire. Cela pourrait remettre en cause, précisément, la justice de proximité, qui est nécessaire.

un pas significatif et clair en faveur des victimes, qui mettent du temps avant de déposer plainte, qui déploient un courage extraordinaire et qui voient leur démarche aboutir à des classements sans suite, parce que les moyens de la justice ne sont pas alignés sur les besoins du terrain.

à voter ?… Le scrutin est clos.

des magistrats. Il nous semble important de renforcer les moyens de la formation des forces de l’ordre et des magistrats au traitement spécifique des affaires sexistes et sexuelles. En Espagne, où les juges et les En Espagne, où les juges et les magistrats reçoivent une formation spécialisée sur les violences de genre, les féminicides ont diminué de 25 % sur vingt ans, grâce à une approche intégrée et beaucoup plus rigoureuse.

Un nouveau parcours de formation a été créé en 2024 pour les magistrats. Le cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales permet une spécialisation sur deux ans.

tend à créer 1 000 postes d’attachés de justice, qui sont nouvellement intégrés dans l’organisation judiciaire française et dont les missions incluent l’assistance aux magistrats, la rédaction de décisions et la gestion de contentieux. Compte tenu de la surcharge chronique des magistrats, il nous semble que les attachés de justice pourraient absorber une partie des tâches administratives et préparatoires, libérant ainsi les magistrats pour les questions plus complexes. Par ailleurs, les attachés de justice bénéficient de passerelles vers l’ENM après trois ans d’expérience, ce qui en fait une source potentielle de magistrats complémentaires. Pour ces différentes raisons, il nous semble que la création de 1 000 postes supplémentaires d’attachés de justice permettrait de contribuer significativement à l’amélioration du système judiciaire français, en répondant notamment à la surcharge des magistrats. Quel est l’avis de la commission ? Je le rappelle,

adoptés permettent d’accroître ces engagements et de nous rapprocher des objectifs de la programmation, notamment s’agissant des recrutements et de l’attractivité des métiers. Des efforts importants ont déjà été consentis. Les effectifs des catégories A et des magistrats ont connu ces dernières années une hausse rapide, ce qui traduit le plan de recrutement pour les magistrats, de 9,1 % en cinq ans, mais aussi la revalorisation des statuts des personnels. L’augmentation des emplois travaillés du personnel d’encadrement de catégorie A, en hausse de 23,6 % pour la seule année 2025, illustre le passage de certains greffiers de la catégorie B à la catégorie A, en application de la réforme statutaire des greffes. Ces réformes portent leurs fruits. D’ailleurs, au cours des auditions que j’ai menées, on m’a signalé que le nombre de candidats au dernier concours de greffier avait été deux fois plus élevé qu’au concours précédent. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

mois de septembre de cette année, le tribunal judiciaire comptait 16 magistrats du siège et la promesse avait été faite d’une dix septième arrivée. Or deux juges aux affaires familiales

2025. En parallèle, le nombre de magistrats localisés au parquet n’a pas évolué depuis vingt et un ans. Nous sommes à 1,37 magistrat pour 100 000 habitants. C’est le parquet le plus faiblement doté de la cour d’appel de Rennes. La moyenne nationale est à 3,2 et la médiane européenne à 11,2.

la commission. Je suis conscient des efforts qu’il faut poursuivre en direction de la justice.

Vous le savez, en France, un enfant est tué tous les cinq jours et 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Malgré cela, nous n’avons pas assez de juges ! Chaque magistrat doit

supplémentaires. C’est un investissement, certes, significatif, mais qui nous paraît soutenable dans le cadre des 10 000 recrutements prévus par le ministère de la justice. Cela permettrait de

lorsque le déplacement est possible dans ce délai, il implique une disponibilité particulièrement longue de l’avocat concerné, ce qui rend la mise en œuvre de ce droit particulièrement complexe.

Toutefois, il est illusoire d’imaginer tout régler à court terme par un mécanisme de régulation carcérale. D’ailleurs, si le comité des États généraux de la justice aborde cette piste, c’est davantage dans une perspective de moyen terme, avec un double mécanisme de seuil d’alerte et de seuil critique. De plus, il n’y a pas pas de consensus aujourd’hui sur la forme que devrait prendre un tel mécanisme de régulation, et ce n’est pas en créant un programme que nous pourrons résoudre cette difficulté. Votre proposition nous permet cependant d’interroger le Gouvernement sur les suites qu’il entend donner à cette réflexion. En conséquence, je sollicite le retrait

Le centre pénitentiaire de Majicavo illustre une réalité alarmante : on y dénombre 620 détenus pour 278 places, soit un taux d’occupation de 252 %. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils révèlent une véritable urgence humanitaire. En mars 2022, le garde des sceaux avait promis un nouvel établissement. Eh bien, deux ans et demi plus tard, le chantier n’a toujours pas avancé d’un centimètre

mais ses auteurs souhaitent avant tout alerter sur la situation dans ce département. Les émeutes survenues le 28 septembre dernier ont été particulièrement éprouvantes pour le personnel de l’établissement, qui est l’un des plus surpeuplés de France. de France. La création d’un second établissement avait été annoncée, me semble t il, par le précédent garde des sceaux. Je ne suis pas sûr que le frein principal soit lié au financement : la construction d’un établissement pénitentiaire nécessite de trouver un site adapté en matière de sécurité et d’accès, mais aussi de prendre en compte les oppositions locales.

au regard notamment du relief très accidenté de l’île, de difficultés d’accès en dehors des agglomérations et d’une desserte limitée en réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement. Aussi, monsieur le sénateur, je vous

Cet amendement d’appel vise à adapter les prisons aux détenus en situation de handicap. L’Observatoire international des prisons (OIP) note que si deux arrêtés fixent des quotas de cellules pour personnes à mobilité réduite, selon un état des lieux, moins d’un établissement sur deux en est doté. La mise aux normes des établissements est souvent tardive, voire inexistante. L’OIP a documenté à plusieurs reprises des atteintes aux droits des personnes incarcérées en situation de Par exemple, on apprend que, dans une prison, en raison du dysfonctionnement fréquent de l’ascenseur depuis plusieurs années, les personnes handicapées restent confinées au troisième étage, devenu en quelque sorte une prison dans la prison. Un détenu témoigne : « Je me retrouve à l’écart des autres. Au dernier parloir, ma famille venue de loin n’a pas été prévenue que l’ascenseur était de nouveau en panne. Ils ont fait le trajet pour rien. » Dans une autre prison, l’administration pénitentiaire avait proposé à un détenu d’être porté dans les escaliers par deux détenus auxiliaires, tout en leur faisant signer tout de même une décharge de responsabilité en cas d’accident. Rappelons que, dans un arrêt de 2006, la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que « la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule par ses propres moyens » constituait un « traitement dégradant

L’aide aux victimes, notamment aux femmes victimes de violences, nécessite des moyens à la hauteur, ainsi que le Gouvernement s’y est engagé le 25 novembre dernier lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la mission gouvernementale sur la soumission chimique que je mène avec ma collègue députée Sandrine Josso

du Gouvernement ? Le budget qui est présenté comporte déjà une hausse des crédits dédiés à l’aide aux victimes. J’ai d’ailleurs eu un échange cette semaine avec les responsables de France Victimes. Je vous indique que la compensation du coût de la revalorisation salariale dite Ségur est prévue dans le cadre de l’amendement n° II 900, qui sera présenté par le Gouvernement. Madame

Il existe un poste de coordonnateur secrétaire général au sein du conseil départemental de l’accès au droit et de la médiation (CDAD) de Mayotte. Ce poste est actuellement pourvu. Il convient de noter, par ailleurs, qu’une nouvelle présidente du CDAD a pris ses fonctions en septembre 2024. lors de l’exercice précédent, l’action du CDAD de Mayotte s’est déployée cette année dans trois axes majeurs : les actions à destination du public, les actions d’information et de formation et le développement d’outils de communication. Si les diverses crises ont entraîné un ralentissement

pour la numérisation des procédures judiciaires. Les investissements consacrés aux outils numériques ont été insuffisants ou mal gérés, marqués par des priorités fluctuantes et des externalisations excessives. Cela limite la modernisation de notre des processus judiciaires. En guise de comparaison, des pays comme l’Estonie ou les Pays Bas, qui sont souvent cités comme étant des leaders dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la justice, disposent de plateformes intégrées pour la gestion électronique des dossiers, l’accès aux jugements en ligne et la communication numérique sécurisée. Ces systèmes améliorent les délais de traitement et la transparence. Le manque de formation des personnels judiciaires freine l’adoption des outils numériques. Un effort est nécessaire pour former les utilisateurs aux nouveaux systèmes et éviter les résistances institutionnelles. En outre, les tribunaux manquent souvent

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice » figurant à l’état B. Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite. Je vous rappelle que la commission des finances est favorable à l’adoption des crédits de cette mission. Je mets aux voix ces crédits, modifiés. Nous

s’appuierait uniquement sur le nombre de mesures de réparation des dommages causés prononcées ne constituerait pas un bon indicateur de performance. Son interprétation serait en effet très difficile, dans la mesure où la précision des données recueillies dépendrait de la nature de l’action engagée, mais également du

Quel que soit le sort qui sera réservé à la motion de censure qui sera débattue demain à l’Assemblée nationale, je sais que le ministère de la justice pourra toujours